La séance est ouverte, le compte rendu analytique de la présidente de séance a été distribué, il n'y a pas d'observation, donc le procès verbal est adoptée sous les réserves d'usage j'informe le Sénat que des candidatures ont été publiés pour siéger au sein d'une part de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance du 19 janvier 2017 relatives à la profession de physicien médical et l'ordonnance du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé et sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance du 27 avril 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives. Relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé. Et d'autre part de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance. Du 3 mai Du 3 mai 2017 portant création de l'établissement public Paris La Défense, les candidatures seront ratifiées si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévue par notre règlement. J'informe également le Sénat que les candidatures pour siéger au sein de plusieurs organisme extraparlementaire ont été publiés ces candidatures seront ratifiées si la présidence n'a pas reçu l'opposition dans le délai d'une heure prévue par notre règlement. Maintenant, l'heure du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances adoptées par l'Assemblée nationale pour 2018 : nous poursuivons l'examen au sein de la seconde partie du projet de loi de finances des différentes missions. Le Sénat va examiner les crédits d'émission, pouvoirs publics conseillés et contrôle de l'État et direction de l'action du gouvernement et du budget annexe publications officielles et information administrative. la parole est à madame Christine Lavarde en remplacement de Monsieur Albéric de Montgolfier, rapporteur spécial de la commission des finances pour la mission, pouvoirs publics. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, effectivement je remplace matin Albéric de Montgolfier, rapporteur spécial de cette mission qui est retenu pour une réunion relative à la conférence nationale des territoires, il a souhaité vous adresser ses mots, les pouvoirs publics participent pleinement à l'effort de redressement des comptes publics, comme en attestent les montants des crédits demandés dans le cadre du projet de loi de finances que nous discutons actuellement pour l'exercice 2018 les crédits s'élève à 991007 millions d'euros en stabilité presque parfaite par rapport à 2017, soit exactement, plus 0,0 dans le détail cette évolution recouvre une stabilisation des dotations de l'État aux assemblées parlementaires et à la Cour de justice de la République, une progression de salles à la présidence de la République et une diminution des crédits du Conseil constitutionnel, commençons par la présidence de la République dont la dotation est porté de 100 millions d'euros en 2017 à 103 millions d'euros l'année prochaine, cette augmentation de 3 qui succède à 3 exercices de reconduction à l'identique de la dotation est justifié par une mise à niveau des équipements destinés à assurer la sécurité des personnes et des biens, les charges de personnel progresse de 1,6 millions d'euros, soit plus 2 2 3 pourcent en raison du renforcement des effectifs de sécurité autour du chef de l'État, les effectifs affectés à des missions de sécurité représentant représentant près du tiers de l'ensemble des personnels de la présidence, venons-en à présent autant aux 2 assemblées dans le cadre du projet de loi de finances pour 2018 les dotations versées à l'Assemblée nationale et au Sénat, s'élève à 841,5 millions d'euros, montant inchangé depuis la loi de finances pour 2012, cette stabilisation en euros courants des dotations des 2 chambres est associée à la réalisation d'efforts en dépenses qui permettent d'absorber en partie la hausse tendancielle de leur charge les dépenses de l'Assemblée nationale reculerait de 34,7 millions d'euros en 2018, soit une baisse de 5,9 pourcent la dotation de l'État est maintenu à 517,89 millions d'euros, un prélèvement sur les disponibilités financières de l'Assemblée nationale, d'un montant de près de 28 virgule 5 millions d'euros, contre 62,8 millions d'euros en 2017 permettant d'équilibrer le budget, la dotation de l'État au Sénat, au titre de l'exercice 2018 demeurent également au même niveau depuis 2012 soit 323 58 millions d'euros, illustrant la poursuite des efforts engagés depuis 2008, les dépenses du Sénat diminuerait sensiblement en 2018 en marquant un recul de près de 12 millions d'euros, soit 3,29 pourcent comme l'Assemblée nationale, le Sénat équilibreraient son budget 2018 par un prélèvement sur ces disponibilités financières d'un montant de 22,2 millions d'euros pour ce qui est de la Chaîne parlementaire, le projet de budget pour 2018 de LCP Assemblée nationale prévoit une dotation de 16,64 millions d'euros, identique à celle de 2017 la dotation demandée par Public Sénat est en diminution de 1,1 pourcent en 2018 à 18,5 0 5 1000000 d'euros, ces dotations sont conformes à la trajectoire définie par le contrat d'objectifs et de moyens signé en décembre 2015 pour la période 2016, 2018 la dotation demandée par le Conseil constitutionnel au titre de 2018 et quant à elle, en baisse de 1 virgule 90 8 millions d'euros et s'élève à 11,7 millions d'euros, la différence correspond au montant prévu pour 2017 pour financer les dépenses relatives à l'élection présidentielle, la baisse de 120000 euros, des dépenses de fonctionnement, équilibre, la hausse du même montant des dépenses d'investissements consacrés à des équipements informatiques et des travaux de restauration de différents espaces alors que la réforme constitutionnelle de Dominique avec institution de la question prioritaire de constitutionnalité a conduit à 2 à une forte hausse de l'activité de la juridiction, le budget du Conseil constitutionnel pour 2018 est inférieur de près de 1 de 6 pourcent à la dotation accordée en 2009, j'en viens pour terminer à la Cour de justice de la République à titre de rappel, conformément à l'article 68, tiré de la Constitution, la Cour est compétente pour juger les membres du gouvernement, au titre des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, le budget prévisionnel de la Cour de justice de la République s'élève à 861500 euros, soit un niveau identique à celui prévu depuis 2015, je vous rappelle que le président de la République s'exprimant le 3 juillet 2017 devant le Congrès, a indiqué sa volonté de voir supprimer cette institution en conclusion, la commission des finances vous propose l'adoption sans modification des crédits de la mission, pouvoirs publics, je vous remercie. Merci. Donc, la parole est maintenant à monsieur Didier Rambaud, rapporteur spécial de la commission des finances pour la mission conseil et le contrôle de l'État. Si le président, Monsieur le Ministre Madame messieurs les rapporteurs mis chers collègues, cette mission, contrôle de l'État, regroupe les crédits de plusieurs institutions, dont le Conseil d'État et les juridictions administratives, la Cour des comptes et les juridictions financières, le Conseil économique, social et environnemental et le Haut conseil des finances publiques, le budget de cette mission s'élève à 665 millions d'euros en crédit de paiement pour 2018 compte tenu de l'amendement de majoration de 2,1 millions d'euros, adopté en seconde délibération à l'Assemblée nationale, le montant des crédits alloués au Conseil d'État et aux autres juridictions administratives demeure le plus élevé de la mission avec 406,7 millions d'euros les juridictions administratives concentre par ailleurs cette année l'ensemble des créations d'emplois de la mission parmi les 54 emplois créés 51 sont affectés à la Cour nationale du droit d'asile, laquelle doit faire face à une augmentation continue du contentieux de l'asile, plus particulièrement en 2017 avec une progression de 30 les 3 derniers emplois créés sont issus des juridictions judiciaires afin de pourvoir les postes de magistrats de la commission du contentieux du stade du stationnement payant cette commission qui verra le jour dès janvier 2018 aura en elle-même peu d'incidence sur le budget du programme ces moyens étant principalement retracé dans la mission administration générale et territoriale de l'État, cependant, le Conseil d'État demeure juge de cassation de discussions de cette commission et pourrait donc connaître une augmentation des affaires en 30 ans s'était vendu alité préoccupante au regard de l'accroissement global du contentieux administratif, lequel n'est pas nous, pas non plus les cours administratives d'appel ou les ou les tribunaux administratifs, les contentieux de masse occupent toujours une part importante des affaires entrants tels que le contentieux du droit au logement opposable 7 pourcent du contentieux, Total et sur lequel je suis assez circonspect monsieur Ministre l'ampleur des moyens mis en oeuvre pour le traitement du contentieux du droit au logement opposable semble très importante au regard du peu qu'on les procédures, en effet enfin veiller à ce que les moyens des juridictions administratives suffisent pour qu'elles respectent leur objectif de délits et de jugement raisonnables, ce qui semble, pour 2018 le budget du Conseil économique, social et environnemental, c'est à 40 millions d'euros en 2018 cette assemblée des corps intermédiaires, poursuit sa modernisation engagée depuis 2015 le CESE cherche en effet à réaffirmer sa mission consultative en produisant des avis en lien avec d'autres institutions comme la Cour des comptes ou le défenseur des droits ou en se saisissant de sujet recueillant un grand nombre de pétitionnaires sur Internet, ce projet de modernisation du CESE pourrait être prolongé avec la réforme annoncée par le président de la République en juillet dernier, devant le Congrès, peut-être pourriez-vous, Monsieur le Ministre, nous en dire un peu plus sur le calendrier et les contours de cette réforme peut dévolution sont attendues sur le programme, la Cour des comptes et autres jurés juridictions financières les crédits augmentent peu pour 2018 il y atteindront 218 millions d'euros, je m'interroge cependant sur la possibilité pour ce programme d'accueillir en son sein les crédits du Haut Conseil des finances publiques sous la forme d'une action ces crédits sont depuis 2014 présenté dans un programme à part, alors que les moyens consacrés au fonctionnement du Haut Conseil son dossier, issu de la Cour des comptes, ce programme ayant été créé par une loi organique, il faudrait donc aucune modification par ce même canal interviennent aussi, pensez-vous, Monsieur le Ministre, qu'une telle modification pourrait être à l'ordre du jour, alors où on nous parlons de plus en plus de réviser notre procédure budgétaire en conclusion Monsieur le président, Monsieur le Monsieur, le ministre mais, chers collègues, la commission des finances propose d'adopter les crédits de cette mission. Merci donc la parole est maintenant à monsieur Bernard Delcros, en remplacement de Monsieur Michel Kahn bête, rapporteur spécial de la commission des finances pour la mission, direction de l'action du gouvernement.

Monsieur le président Monsieur Ministre, chers collègues, en effet, Michel canevas été retenu aujourd'hui à Rennes, il m'a donc sollicité pour présenter sa mission ce que je fais évidemment avec plaisir en 2018 et les crédits de paiement de la mission, direction de l'action du gouvernement sont légèrement inférieurs à 1,5 milliard d'euros, il relève de 3 programmes le programme 129 coordination du travail gouvernemental, le programme 308 assurant le financement de 11, autorité administrative indépendante et le programme 333 finançant le fonctionnement d'une partie de l'administration déconcentrée de l'État, le budget stable à périmètre constant des mesures périmètre pour 14 millions d'euros correspondent notamment à la mutualisation à laquelle participe le Commissariat général à l'égalité des territoires, dans le cas de l'installation de 15, service dépendant du 1er mini-sur le site de Ségur Fontenoy ce projet au coût total de 370 millions d'euros, cancer, les locaux de l'ancien ministère de la mer et une partie de l'ancien ministère de la Santé, le défenseur des droits, et la CNIL s'y sont installées l'année dernière, réalisant ainsi une économie annuelle d'environ un 1000000 d'euros en loyer et c'est aujourd'hui le tour des différents services dépendant du 1er ministre à périmètre courant les dépenses d'intervention augmente de 7 millions d'euros, 4 millions sont prévus pour l'indemnisation des victimes des essais nucléaires et 2,7 millions. Pour la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et la haine anti-LGBT 18 créations d'emplois sont prévues, essentiellement dans le programme de coordination du travail gouvernemental, qui compte 700 millions d'euros de crédits consacrés pour moitié au secrétariat général de la défense et de sécurité nationale. Priorité a été donnée à la lutte contre le terrorisme et au développement de renseignement, les crédits dévolus à ce secrétariat général augmente, notamment au profit de l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information qui agit pour assurer la sécurité informatique de l'État et des opérateurs d'importance vitale les moyens augmentent aussi pour le Groupement interministériel de contrôle chargé des opérations d'écoute sur le territoire, or écoutes judiciaires les crédits des autorités administratives indépendantes sont relativement maîtrisé, un peu moins de 100 millions d'euros, donc 40 pourcent 2 d'entre le 11, autorité administrative obtiennent des crédits supplémentaires pour faire face à une augmentation de leur activité, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dans la charge de travail s'est accrue et la commission du secret de la défense nationale, le regroupement dans ai parlé permet une réelle mutualisation, notamment sur le plan de la sécurité et des moyens techniques, en particulier de la téléphonie, cela devrait permettre de réaliser des économies en dépenses de fonctionnement, à hauteur de 7 millions d'euros par an d'ici 2022. Il permettra également de céder du Patrimoine immobilier dont la valeur est estimée à environ 160 millions d'euros, enfin en ce qui concerne le programme moyens mutualisés, des administrations déconcentrées Michel Canivet propose rappelle que les systèmes d'information de l'État sans gérés par les services interministériel départementaux des systèmes d'information et de communication qui regroupe 1200 agents responsables des parcs informatiques sur le territoire. Il note toutefois que le fait que les personnels et des statuts différents et soient encore attaché à plusieurs ministères, des problèmes de fonctionnement et qui serait sans doute plus efficace de les doter d'un statut unique et qui soit véritablement rattaché aux services du 1er ministre. Pour le budget annexe 180 millions d'euros sont prévus pour financer la direction de l'information légale et administrative qui bulle publie notamment le Journal officiel, avec des recettes qui couvre les dépenses sa direction participe à la transformation numérique de l'État et gère en particulier les site Legifrance et service public. Michèle Khan, constate avec satisfaction les efforts de gestion de la dit la accentuant une évolution forte vers le numérique, effectuant une maîtrise des crédits par la réduction des moyens humains, il souligne la nécessité de poursuivre les mesures de départs anticipés à la retraite dans la coopérative datant de 2 siècles qui assuré les éditions papier pour le compte de la ainsi notre collègue, comme la commission des finances propose d'adopter les crédits de la mission et du budget annexe, je vous remercie. Merci donc la parole est maintenant à monsieur Olivier Cadic, rapporteur pour Abid, de la commission des Affaires étrangères de la Défense et des forces armées pour le programme, coordination du travail gouvernemental pour 3 minutes.

il faut s'en réjouir car il porte les moyens de services indispensables à la politique de défense et de sécurité de notre pays, c'est pourquoi la commission des Affaires étrangères de la Défense et des forces armées a donné à l'unanimité un avis favorable à l'adoption des crédits de cette mission. Je concentre mon intervention sur les crédits attribués à la cybersécurité. Premières observations si l'Autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information représente 60 pourcent des effectifs du programme et le tiers des crédits, or, titre de l'action de pourtant, ils ne font pas l'objet d'une présentation distinctes dans le programme annuel de performance, ce serait un moyen de distinguer les efforts en matière de cybersécurité et les moyens dévolus aux autres missions du SPD la commission demande que l'ainsi soit à la Star du GIC, considéré comme une unité opérationnelle et que la maquette de présentation du programme soit modifié dans ce sens. 2ème observation tous les indicateurs sont au rouge en matière de cybermenaces Lance il va poursuit sa montée en puissance et c'est une bonne chose, mais pourquoi ralentir le rythme de moitié, de 50 créations d'emplois par an à 25 et attend 2022 pour atteindre le niveau optimal des besoins exprimés par l'agence. Ces missions vont s'accroître tant dans le cadre de la mise en Oeuvres de la directrice, que des mesures qui seront issus, on peut pronostiquer de la revue de stratégie sidère actuellement menée par le SGDN ne peut donc accélérer la montée en puissance, les problèmes de recrutement qu'a connu l'homme s'il semble largement résolue mais il faudra demeurer vigilants car le vivier des spécialistes recrue tables et faible et la concurrence est notre commission estime qu'au-delà de la politique de labellisation une politique active de développement de filières de formation initiale par une application plus forte du ministère de la recherche de l'enseignement supérieur et des partenaires économiques est indispensable, le 1er ministre entend-il avancer sur ce terrain. Dernière observation, 3 ans après la publication de la circulaire du 1er Ministre exposant la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État et fixant des règles de protection le niveau effectif de conformité des systèmes d'information de l'État tarde atteint les cibles en adéquation avec les enjeux, le comblement du retard souffrent de l'insuffisance des moyens organisationnels et budgétaires, le service interministériel de supervision confia à Lance, il se heurte à des contraintes techniques et d'organisation qui ne permet pas toujours de déployer ses sondes sur les réseaux dans les conditions adéquates ni de recueillir toutes les informations nécessaires pour assurer, c'est qu'une détection optimale cette situation reste insatisfaisante et la Commission s'en inquiète, elle demande qu'une évaluation soit conduite par un corps d'inspection pour identifier les difficultés et proposer un plan d'action, elle souhaite également que soient étudiés sur les plans juridique et technique les moyens pour le MC de contraindre et d'imposer ses préconisations aux directions des systèmes d'information, des ministères, je vous remercie. Merci, la parole est maintenant à monsieur Rachel Mazuy, rapporteur pour avis de la commission des Affaires étrangères de la Défense et des forces armées pour le programme, coordination du travail gouvernemental. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, si la commission des Affaires étrangères de la Défense et des forces armées a donné un avis favorable à l'adoption des crédits de cette mission, c'est parce que les crédits de l'action 2 du programme 129 coordination de la sécurité de la Défense. Placé sous la responsabilité du secrétaire général pour la défense et secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, connaissent une légère augmentation dans un budget il est vrai, contraint, donc c'est une bonne nouvelle, cette action porte les crédits de nombreux organismes dont, bien sûr, le secrétaire général de la défense nationale, mais aussi l'Agence nationale sécurité dont vient de parler donc Lake Olivier Cadic cap. cap. Groupement interministériel de contrôle et les instituts de formation, que ce soit celui de la Défense nationale ou celui de la sécurité et la justice, donc mes observations porteront sur certains d'entre eux, premières observations, le Groupement interministériel de contrôle J. qu'est devenu le pivot inter- ministériel de gestion de l'ensemble des techniques de renseignement. L'usage de nouvelles techniques, mais surtout la lutte contre le terrorisme entraînante Nater signification significative significative de son activité. Il doit, en conséquence, poursuit sa transformation et sa montée en puissance 11 schéma d'emplois a été revu à la hausse et ses effectifs devraient atteindre 243 équivalents temps plein en 2020, le processus se déroule très normalement. L'effort donc budgétaire est maintenu notre commission avec attirer l'attention du. 1er mini-sur la nécessité de veiller au bon mentionnant du pour une mise en oeuvre 15 de la loi. Nous saluons s'était formés, nous réitérons cet appel à la vigilance. Notamment sur le volet investissement car logique doit équiper ses infrastructures pour accueillir ces personnels actuellement il y a un problème immobilier. Et les exploitants des services tout en continuant à développer les systèmes qui assure conservation et traçabilité des données 2ème observation la diminution si légère soit-elle des fonds spéciaux apprenait justement sensible. En 2017 et reste préoccupante, leur progression devrait accompagner la montée en. Puissance des services de renseignement fortement sollicités, vous vous en doutez, dans le cas de la lutte contre le terrorisme, c'est une recommandation formulée par la commission parlementaire de vérification des fonds spéciaux, donc je crois que la remarque est d'importance pouvez-vous en conséquence nous assurer que l'exercice 2018 constituera une sainte interruption conjoncturel. Dans le processus de sa sécurisation de ces crédits et que l'objectif demeure bien de fixer la dotation à hauteur des moyens nécessaires et prévisible des services 3ème et dernière observation. Les subventions Dallas destinée aux 2 institutions maintenu à hauteur de 13,8 millions après plusieurs années de diminution, ceci devrait, de notre point de vue constituer un choc. Minimum permettant le développement de leurs activités, notamment celles susceptibles de produire des ressources propres toutefois le plafonnement des emplois constitue un frein à la réalisation de cet objectif. Un assouplissement me paraît nécessaire, est-il envisageable. La mutualisation des moyens, et le développement des synergies entre les 2 établissements est désormais installé. Complètement réalisé, vous le savez, sur le site de l'école militaire et c'est donc un objectif à part faire enfin. Nous saluons la démarche de l'institut sécurité je justice qui aura mené de front en 2017, la rédaction d'un nouveau plan stratégique et la négociation dont contrat d'objectifs et de performance avec l'État. Mais nous nous étonnons du retard pris dans la rédaction du contrat d'objectifs et de performance Peyrefitte lors de la relations de défense quand, et j'en ai fini sera-t-il soumis au conseil d'administration. La parole est maintenant à madame Chantal de Seine, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales pour la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, au sein de la mission Direction de l'action du gouvernement, la commission des affaires sociales examine le budget et l'activité de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives cas chargé de l'élaboration et du pilotage de la politique gouvernementale dans ce domaine, elle a émis un avis favorable à l'adoption de ces crédits qui s'élèveront à 17,8 millions d'euros l'an prochain, tout en regrettant que leur diminution qui a débuté en 2013 se poursuivent en effet les nombreux défis auxquels la France soit faire face en matière d'addictions justifierait d'y consacrer des moyens bien plus importants à la veille de l'élaboration de la prochaine stratégie pluriannuelle gouvernementale, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur 3 points, il convient tout d'abord de ne pas répéter les erreurs du plan 2013, 2017 et de ceux qui l'ont précédé, il constituait un catalogue de mesures assez hétéroclite, sur lesquels étaient saupoudrer des ressources limitées, la multiplication des initiatives n'est pas synonyme d'efficacité mais souligne l'incapacité de la puissance publique à identifier les enjeux principaux et à trouver les moyens d'y répondre, il est surtout urgent de réformer dès l'an prochain la réponse pénale à l'usage simple des stupéfiants depuis 1970 celui-ci c'est est puni d'un an de retrouver zone nom et de 3750 euros d'amende jamais appliquée cette peine a perdu tout caractère dissuasif, la levée de cet interdit qui reste pleinement justifié par des considérations sanitaires, sociales et d'ordre public n'est ni souhaitable, ni envisageable toutefois l'amélioration de l'efficacité de l'action pénale est indispensable, alors que les tribunaux et les services de police sont fortement mobilisés par ce contentieux de masse longtemps controversée, la contre-contravention n'a livré à Sion de l'usage fait désormais consensus quel dommage que le gouvernement s'y soit opposés à 2 reprises, lorsque le Sénat le proposait en 2011 et en 2015 le traitement de l'infraction serait grandement simplifiée et accélérée en infligeant une sanction pécuniaire immédiate dont le montant reste à déterminer mais devrait être suffisamment dissuasive et proportionnée à l'infraction commise le caractère virtuel de la sanction actuelle disparaîtrait l'impact en serait d'autant plus fort chez les jeunes, chez qui il faut absolument faire reconduit, faire reculer les conduites à risque, enfin, la commission a particulièrement insisté sur la nécessité de mieux prendre en contre les outre-mer, elle souhaite qu'en préparation de la prochaine stratégie gouvernementale soit conduite une grande étude sur les phénomènes s'addictif dans les départements et collectivités d'outre-mer, sur la base de ces résultats, le dispositif de prise en charge des addictions devra être adaptée aux spécificités de ces territoires, je vous remercie. Merci. Si cher collègue, la parole est maintenant à monsieur Jean-Pierre Sueur, rapporteur pour avis de la commission des lois pour la mission, pouvoirs publics. Et toujours pour 3 minutes. a un monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, donc nous sommes au régime 3 minutes. 3 minutes, finalement, c'est assez peu, je pense que certains pensent d'ailleurs que moi, il y a du débat parlementaire et moins de temps, mieux c'est, finalement, et quand on aime le Parlement, on rêve de l'époque pour Robert Badinter, multiplié par 2 son temps sans qu'aucun président de séance l'interrompre. La force du débat, c'est quelque chose qui n'est pas toujours déterminé, mes chers collègues par le chronomètre bien alors ce budget il y a d'abord l'Élysée, la présidence de la République

et je rappelle que, en 2012, il était de 109 millions d'euros, donc vous voyez mes chers collègues, que nous sommes passés en 2012, 17. De 109 à 100 millions d'euros, donc je rends hommage au président François Hollande qui a fait preuve. D'une vertu d'une maîtrise des finances qui doit être salué alors vous me direz, il y a une augmentation de 3 millions d'euros cette année, hé bien je vais vous dire qu'avec la commission des lois, mes chers collègues, je la soutiens, pourquoi, parce que cette augmentation et s'explique exclusivement. Par des questions de sécurité qui sont dire ils mentent, il est très important que les contacts entre l'Élysée et l'ensemble des chefs d'État étrangers soient sécurisés, qu'en tout lieu du globe, le chef de l'État puisse avoir des relations avec les forces stratégiques avec les armées, et vous savez qu'aujourd'hui il y a une guerre du cryptage du décryptage, qui est considérable, au niveau de la planète et qu'à cet égard. Ce qui a été. Pris comme décision, et qui figure dans le rapport m'apparaît absolument responsable et nécessaire, c'est pourquoi nous soutenons le budget de l'Élysée, avec cette augmentation et pour ces raisons, est entendu que dans d'autres domaines, la maîtrise des dépenses se poursuit pour ce qui est des assemblées parlementaires, hé bien le chiffre reste stable. En francs courants, eu égard au fait que chaque assemblée doit faire appel à ce qu'on appelle disponibilité, c'est-à-dire aux réserves, ce qui n'est pas une solution pérenne pour ce qui est du Conseil constitutionnel. Comme cela a déjà été dit Madame la rapporteur général, hé bien, le Conseil constitutionnel, un budget pratiquement constant. Par rapport à l'exercice antépénultième pourquoi hé bien parce que cette année a été marquée par 3 sélections nationales, l'élection présidentielle élections sénatoriales, élections législatives, ce qui a entraîné. Un coût supplémentaire que l'on ne retrouve pas au cours de l'année 2018. Le président du Conseil constitutionnel a développé une action pour. Les relations internationales, notamment sur le plan de la francophonie, des relations avec l'Allemagne, la cour constitutionnelle d'Allemagne et aussi avec les pays de l'Europe du Sud, nous soutenons cela ainsi que tous les efforts pour mieux faire connaître l'action du Conseil constitutionnel et l'accès aux droits, notamment auprès des jeunes et le droit auprès des jeunes, mais nous insistons sur le fait que cela doit s'inscrire dans le respect de la maîtrise des dépenses, enfin, Monsieur le Président, pour ce qui est de la Cour de justice de la République. Eh bien, j'espère que bientôt, nous n'en parlerons plus. Parce qu'on aura trouvé un autre dispositif qui sera meilleur. Et j'ajoute, à titre accessoire que le coût des locaux restent importants pour cette institution mais, chers collègues, je n'est dépassé que très modérément. Et trop modérément le temps qui m'était impartie et je comprends dans ces circonstances, l'indulgence de monsieur le président je vous remercie. Merci monsieur maire. Si monsieur monsieur Sueur un très léger dépassement en valeur absolue, très forts dépassements pourcentage mais bon, tout est relatif, donc la parole est maintenant à monsieur Patrick Kanner, rapporteur pour avis de la commission des lois pour la mission, conseil et contrôle de l'État. Merci, Monsieur le 1er président juste à vous serez aussi tolérant avec moi, mais je vous rassure, mon discours est écrit ce que c'est même plus simple garder son temps de parole Monsieur le Ministre, Mesdames et messieurs les rapporteurs mais chers collègues pour l'exercice 2018 les juridictions administratives et les juridictions financières bénéfice il faut le constater d'une hausse de leur budget, je vous invite cependant à ne pas vous arrêter aux apparences qui pourrait laisser penser que ces juridictions jouissent de situations privilégiée dans le contexte de rigueur budgétaire que chacun d'entre nous peut connaître les crédits supplémentaires alloués aux juridictions administratives sont en réalité destinées essentiellement et cela été dit tout à l'heure par le rapporteur spécial à la Cour nationale du droit d'asile, qui est confrontée à une progression importante pour ne pas dire exponentielle du nombre de faire entrer cette augmentation des effectifs pourraient déjà être pourtant insuffisante car les 51 nouveaux emplois fléchés permettent la création, ce qui est bien bien de 2 chambres, soit une capacité de traitement de 7000 affaires par an, mais la présidente de la Cour nationale du droit d'asile que j'ai rencontrés lundi dernier, me disait que l'estimation pour 2018 serait de 11000 affaires supplémentaires s'agissant des juridictions nitrates et de droit commun, les délais de jugement inférieure à un an affichés cache une réalité toute autre si l'on retire du calcul des procédures d'urgence encadré dans les délais, contraint, CDD en moyenne sont nettement plus long un an 8 mois 22 jours pour les tribunaux administratifs pour faire face à la pression contentieuse, les juridictions nitrates Yves vont engagé de nombreuses réformes de procédure, tant mieux, développement des télé-procédure multiplication des procédures contentieuses à juge unique, par exemple, mesdames et messieurs les sénateurs, il semble difficile d'aller plus loin sans Porter atteinte à la qualité des décisions de justice, la commission des lois vous propose d'autres pistes d'amélioration comme l'engagement une réflexion portant sur le contrôle de l'attribution de l'aide juridictionnelle, dans le prolongement des travaux de la Haute Assemblée sur le redressement de la justice en veillant cependant et je crois que vous y serez sensible à préserver l'accès à la justice des publics socialement les plus fragiles, c'est aussi une autre idée : le renforcement de l'équipe du magistrat en s'aspirant du statut des juristes assistants qui interviennent auprès des juges judiciaire de notre pays, passons aux crédits alloués aux juridictions financières, ils sont à peine suffisants pour leur permettre d'atteindre le plafond d'emplois fixes depuis 2010, alors même que leur mission continue de progresser : elles ont désormais un véritable rôle d'accompagnement des collectivités territoriales, rendant nécessaire l'adaptation de leurs qui alors il serait pertinent de leur permettre de contrôler des politiques locales, thématiques qui font intervenir une pluralité d'entités différentes en conclusion : malgré le volontarisme et le professionnalisme que j'ai pu constater dont font preuve les magistrats, les personnels des juridictions le constat Michard collègues est sans appel : les gisements de productivité à effectifs constants sont épuisés dès lors aucune nouvelle compétence ne devra désormais être attribué sans une évaluation sérieuse de son apathie sur l'activité de ces juridictions et sans l'allocation de moyens suffisants, sous peine de mettre leur fonctionnement en péril et de porter atteinte à la qualité de la justice rendue pour nos concitoyens, au bénéfice, Monsieur le Président de ces observations, mais aussi toute inquiétude, la commission des lois a mis un avis favorable à l'adoption des crédits de programmes conseil d'État et autres juridictions ministre a-t-il et Cour des Comptes et autres juridictions financières, je vous remercie. Monsieur Kanner, la parole est maintenant à monsieur Jean-Yves Leconte, rapporteur pour avis de la commission des lois pour les programmes, coordination du travail gouvernemental et protection des droits et libertés de la mission Direction de l'action du gouvernement je. Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, cette mission taxi, direction de l'action du gouvernement et budget annexe Publications officielles et information administrative regroupe 3 programmes le programme 129 coordination du travail gouvernemental, principalement le secrétaire général à la défense et la sécurité nationale, c'était d'agir du gouvernement le SGE et le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique, le programme 308 importants programme qui regroupe le budget des autorités administratives indépendantes chargées de la protection des droits et libertés enfin le programme 303 moyens mutualisés, des administrations déconcentrées, c'est un budget globalement de 1 milliard 6 d'autorisations d'engagement et un milliard 5 de crédits de paiement, il a été mis en oeuvre mais pro il est proposé, dans un souci de maîtrise des finances publiques et aussi en tirant bénéfice d'un certain nombre de mutualisation avec les effets de l'opération immobilière Ségur Fontenoy où un certain nombre de d'administration se sont progressivement regroupées depuis 2 ans quelques priorités au point de vigilance sur ces programmes d'abord le rôle de l'Agence nationale des sécurités de systèmes d'information intégrés au secrétaire général à la défense et la sécurité nationale l'Annecy

par des cyber attaques et, indirectement, nous avons vu aussi un certain nombre d'entreprises françaises qui ont été impactés, avec des coûts très importants de plusieurs millions d'euros à l'occasion de cette attaque, en Ukraine, donc c'est la raison pour laquelle il est important que nous ayons un budget sérieux sur ce plan-là ne s'qui a besoin de d'attirer un certain nombre de pour compétence a besoin de moyens pour recruter et et et elle a besoin aussi de la reconnaissance et la capacité d'intervenir dans toutes les administrations, j'ai encore avec douleur le senti le rappeler par internet qui n'ont pas été possible pour les Français de l'étranger, cette année, faute d'une sécurité suffisante, donc là, ne s'y est une priorité, à mon sens très importantes pour les années à venir et de son budget est en légère augmentation, le SGA qui aura comme rôle de défendre les positions françaises au moment du Brexit mais aussi qui doit disposer des moyens adaptés aux ambitions de la France pour l'Europe, et en Europe, alors les autorités administratives indépendantes qui sont des contre-pouvoir indispensable dans une société qui demandent de plus en plus de technicité je voudrais rendre ici un hommage particulier à l'c'était qui alors que j'ai voté contre la loi sur le renseignement, il y a quelques années rend crédible les dispositions qui ont été mis en place dans cette loi et qui dispose des moyens pour travailler correctement, la CNIL, qui fera l'objet, l'année prochaine d'une profonde modification avec la mise en oeuvre du nouveau règlement européen sur la protection des données personnelles que nous devrons transposée au début de l'année prochaine, le défenseur des droits essentiels pour lutter contre les 10 que discrimination et qui a comme nouveau rôle maintenant la protection des lanceurs d'alerte, enfin, le contrôleur général des prisons et le CSA enfin monsieur le ministre, en conclusion, je voudrais attirer quand même votre attention sur une préoccupation relative à la réduction des cabinets ministériels, un lien entre les ministres et des administrations, plus Direct, ça peut sembler intéressant sur le plan théorique, et c'est un peu je crois l'idée qui a été développé par le nouvel exécutif mais nous n'avons pas l'impression que ça fonctionne réellement bien aujourd'hui que ce soit dans les contacts avec les élus, mais aussi parfois en ministériel une note que j'ai intégré à mon rapport du directeur de cabinet du 1er Ministre cadre un peu nouveau fonctionnement de l'administration, il y a un peu finalement différent de notre de nos traditions habituels, mais attention à une administration qui évoluerait vers un moindre contrôle politique et un fonctionnement un peu trop sur même ça risque de ne heurter non non non non, notre histoire, mais aussi le contrôle démocratique sur l'administration, alors Monsieur Dini sous ces réserves, la commission des lois a donné un avis favorable à ces crédits et vous demande de veiller à tous ses points au budget des administrations des autorités administratives indépendantes et aussi de bien veiller à ce que le ministre Sion et la réduction des cas ministérielles permettent quand même un fonctionnement de l'État correct, je vous remercie. Merci dans la suite de l'Ain, discussion, je vous rappelle que le temps de parole attribués à chaque groupe pour chaque unité discussion comprend à la fois le temps d'intervention en général et celui de l'explication de vote par ailleurs le gouvernement dispose au total de 10 minutes pour intervenir le dans les interventions générales, la parole est à madame Véronique Guillotin, pour 6 minutes.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre Mesdames, messieurs les rapporteurs, chers collègues, nous sommes réunis, merci, il se réunit aujourd'hui pour examiner les Budgets des 3 missions et un budget annexe l'émission, pouvoirs publics et contrôle de l'État appelleront peu de remarques de ma part, on peut néanmoins noter que si les Budgets du Sénat et de l'Assemblée nationale sont stables, celui de la présidence de la République, progresse de 3 pourcent pour atteindre 103 millions d'euros, alors qu'il stagnait à 100 millions d'euros les années précédentes, bien que cette eau soit justifiée par un renforcement nécessaire de la sécurité et la création de la Task force en même temps je crois aux vertus de l'exemplarité, y compris au plus haut sommet de l'État depuis leur création en 99 les chaînes parlementaires LCP et Public Sénat figure également dans la mission, pouvoirs publics, leur fusion, propice à l'arrêt à la rationalisation est une évolution que nous soutenons, nous accueillons également favorablement la proposition de suppression de la Cour de justice de la République, annoncé par le président en juillet dernier, son budget de 800 61000 euros apparaît excessif au regard du faible nombre de décisions rendues et maintenir une juridiction d'exception pour les membres du gouvernement ne peut plus être aujourd'hui compris par nos concitoyens. Au sein de la mission Direction de l'action du gouvernement, on observe que l'augmentation des effectifs est concentrée sur les organes de sécurité, les autorités administratives indépendantes et les services du secteur de la protection des libéraux dit liberté connaissent cependant une stabilisation, voire une diminution de leurs effectifs, 5 autres ETP de moins pour la défenseur des droits, ce que nous regrettons venons maintenant à la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives la mise des câbles qui conserve des effectifs stables : ces 2 opérateurs le centre interministériel de formation anti-drogue et l'Observatoire français des drogues et toxicomanies conservent aussi leur crédit, nous en sommes satisfaits je vais concentrer mon intervention sur cette mission, la 1000 des cas a pour objectif, grâce à un dispositif transversales, de coordonner les actions à l'échelle nationale, il est question bien sûr ici de budget mais à travers le budget, c'est surtout la situation des addictions en France et son évolution qui nous intéressent tous je crois. La liste des produits concernés, visible sur le site internet de l'ami DK Tabac Alcool, stupéfiants psychoactifs mais le Champ des addictions et plus large et s'étend aux addictions sans produits comme la dépendance aux jeux d'argent, jeux de hasard ou aux écrans, bref, il s'agit surtout d'un problème de comportement que de l'objet de la dépendance, lui-même, je ne reviendrai pas en détail sur le tabac qui a nourri les dettes les débats au cours du PLFSS et dont personne n'ignore plus les effets délétères sur la santé, la mortalité évitable et l'impact des pathologies induites sur les comptes sociaux, malgré les plans gouvernementaux successifs, la situation de la France vis-à-vis du tabac reste préoccupante et il en est de même pour l'alcool, concernant ces 2 substances la France caracole en tête dans le dans le peloton de tête des pays de l'OCDE. La hausse des taxes sur le tabac est inscrite dans le PLFSS 2018, je suis favorable à condition, comme je l'ai dit et comme s'y est engagé Madame la ministre des solidarités et de la santé, qu'elle soit accompagnée de mesures de prévention et de lutte contre la contrebande, parlant du cannabis, quant à lui, qui reste de loin le stupéfiant plus consommer, il est encore trop souvent banalisés, pourtant il est prouvé qu'il est un produit dangereux, responsable de troupes de l'attention de la mémoire baisse de motivation et constitue un risque non négligeable de décompensation de pathologies psychiatriques, il doit rester à mon avis un produit illicite,

ce qui donne un sentiment d'impunité et d'impuissance des pouvoirs publics et les résultats en plus ne sont pas au rendez-vous, la contravention analyse Sion de l'usage, proposition du président de la République, sans pour autant lever l'interdit est un débat qui mérite d'être posée, quelques minutes pour évoquer ces 3 missions, c'est un peu court pour être exhaustif, pour ce qui est de la 1000 écart je vous renvoie à l'excellent rapport détaillé de la sénatrice Chantal de scène de la commission des affaires sociales, que je partage pour l'essentiel, pour conclure, je regrette vraiment les baisses de financement qui se poursuivent dans cette mission, moins 25 pourcent depuis 2012 ans et qui pose la question des moyens alloués face à l'ampleur du phénomène des addictions au vu des enjeux, un Grenelle de la prévention remplacerait avantageusement l'empilement de mesures successives, relevé par la rapporteure

j'invite le gouvernement à moduler, si possible, cette répartition, ce serait un signal fort en faveur de la lutte contre les dépendances, car si les équilibres budgétaires et la sécurité sont importants et nous ne le nions pas la santé de la population, l'est tout autant : plus de prévention, c'est une fine et moins de soins et in fine et des économies à réaliser, je vous remercie. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues permettez-moi d'abord de regretter la fusion de ces 3 missions dans une discussion commune, notamment au regard de l'importance des programmes qui composent qui la composent qui composent, celle de la direction de l'action du gouvernement aux 5 minutes je mettrai donc l'accent que sur certains programmes et feraient l'impasse bien évidemment sur sur sur la mission, pouvoirs publics, aujourd'hui seul avait déjà été dit le Parlement est un peu mis à à la diète, or l'inflation législative et la nouvelle façon envisager de travailler en commission exigée ou exigerait des moyens supplémentaires actuellement les dotations des petits groupes ne permettent pas de toutes les filles de toute évidence, et je sais de quoi je parle, à travail à la hauteur des changements en cours et des exigences constitutionnelles, la question des moyens doit être au centre d'une nécessaire revalorisation du Parlement sur la dotation de la Cour de justice de la République, nous notons que le coût des travaux de cette institution est bien trop élevé, d'autant qu'il s'agit d'une institution sursis comme l'a annoncé le président de la République au congrès de Versailles en juillet dernier, pour notre part, nous soutenons la proposition de renvoi des membres du gouvernement devant les juridictions de droit commun sur la mission conseil contrôle de l'État, on peut saluer l'augmentation du budget pour l'autre programme 165 de la Cour nationale du droit d'asile de 2 millions d'euros sur l'exercice et la création de 51 équivalents temps plein cet effort budgétaire est nécessaire dans le contexte de crise migratoire que nous connaissons bien qu'il soit loin d'être proportionnelle aux 30 pourcent d'augmentation des recours de cette juridiction, en revanche, le programme 126 relatif au Conseil économique, social et environnemental pose question : les missions actuellement attribués à à cette instance justifie-t-elle le budget colossal qui est dédiée à celui-ci et qui est sans cesse abondée nous ne croyons pas une réforme de cette institution semble indispensable, l'idée d'une véritable 3ème chambre citoyenne à émerger, il faut qu'elle mûrisse le programme 340 au conseil des finances publiques, tire les conséquences de l'adoption du pacte de stabilité européen que nous n'avons cessé de dénoncer au groupe CRC l'existence même d'une telle instance quelque que soit son budget pose de sérieuses questions plan du respect des principes démocratiques et de la souveraineté budgétaire du Parlement, enfin sur la mission, direction de l'action du gouvernement, l'augmentation des moyens, des moyens alloués en matière sécuritaire doit nous conduire à nous assurer que dans le même temps, les droits et libertés fondamentales sont bien respectées, c'est ce que révèle avec justesse le rapport de monsieur Leconte mais contrairement à lui, nous pensons que l'équilibre est loin d'être assurée, alors que les effectifs de la et du GIC sont augmentées, dans le même temps que dans le même temps, ne soit pas accordé les quelques ETP qu'aurait souhaité le défenseur des droits, nous le reconnaissons amèrement étant donné l'importance des travaux de cette autorité du programme de protection des droits et libertés de rang constitutionnel qui, rappelons-le, réunit notamment les compétences du médiateur de la République de la Haute autorité de la lutte contre les discriminations et pour l'égalité et du défenseur des enfants, dans le contexte, l'état d'urgence répétés de loi antiterroriste qui a considérablement renforcé les pouvoirs administratifs de l'État, les crédits du défenseur des droits, on est dû être largement renforcé d'autant que chaque nouvelle loi lui confier de plus en plus de missions et donc un Champ d'intervention toujours plus large, or que se passe-t-il au contraire l'activité au siège du défenseur des droits pourraient être affectés en raison de la précarité des emplois de 8 agents qui sont mises à disposition de l'institution par des organismes par notre organisme, ces employes qui n'entrent pas dans le plafond, mais sont rémunérés par le défenseur des droits peuvent en effet prendre fin à tout moment d'autres crédits, aurait dû être renforcée, par exemple, cela été dit, ceux de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et conduite addictive à l'heure où les enjeux en terme de santé publique sont énormes et ce sur l'ensemble de notre territoire se aussi du contrôleur général des lieux de privation de liberté qui s'inquiètent d'une possible régression des droits perçus par certains comme un luxe écrin par exemple une dégradation des droits des étrangers y compris mineurs dans un futur projet de loi relatif à l'immigration, la course au tout sécuritaire dans laquelle se trouve piégé et le gouvernement se traduit dans ce budget et notamment dans le déséquilibre des dotations renforcée pour la sécurité au détriment des lots des droits et des libertés fondamentales, nous ne soutiendrons donc pas les Budgets de ces 3 missions. Merci, la parole est maintenant à Madame Colette Mélot. Toujours pour 5 minutes. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui les crédits dédiés aux mission pouvoirs publics conseillent, contrôle de l'État et direction de l'action du gouvernement ces missions qui touchent au coeur du fonctionnement des institutions républicaines sont stratégiques à plus d'un titre, j'évoquerai tout d'abord la mission, pouvoirs publics, ces crédits n'augmente que de 0 0 8 pourcent entre 2017 et 2018 le budget des 2 assemblées, comme c'est le cas depuis 5 ans 518 millions d'euros pour l'Assemblée nationale et 323 millions pour le Sénat, soit plus de 80 pourcent des crédits de la mission, nous saluons cet effort de modération de la dépense publique qui ne se fait pas au prix d'une qualité de prestation dégradées, je crois d'ailleurs que la qualité et le dévouement des fonctionnaires qui nous accompagne ici au Sénat nous démontrent au quotidien, nous estimons néanmoins que, pour l'avenir, la fin du cumul des mandats et la baisse attendue du nombre de parlementaires ne devront pas mettre en péril les ressources qui nous sont nécessaires pour agir, le Parlement ne pourra exercer la l'ensemble de ses rôles constitutionnel avec rigueur et efficacité que si on lui conserve les moyens de ses attributions en ce qui concerne la mission conseil et contrôle de l'État, nous saluons le rôle fondamental du Haut Conseil des finances publiques du Conseil économique, social et environnemental de la Cour des Comptes et du Conseil d'État dans la définition, le contrôle et l'analyse des politiques publiques, les crédits affectés à ces 4 programmes s'établissent à 680 millions d'euros Anne autorisations d'engagement et 665 millions d'euros en crédit de paiement, cela représente une hausse d'environ 1 pourcent cette progression relativement modéré est encore une continuité avec les lois de finances des années précédentes mais ne reflète pas, à notre sens, l'accroissement des missions dont les juridictions administratives notamment, sont accablés

la Cour nationale du droit d'asile, a également connu ces dernières années une hausse structurelle de son activité due à la croissance du contentieux des étrangers, le gouvernement a identifié ces points de tension mais il répond que de manière modeste, la crise des migrants et l'inscription de nombreuses dispositions de l'état d'urgence dans le droit commun nous semblent au contraire appelé un renforcement en franc et massif de nos institutions juridictionnelles, j'en viens à la mission Direction de l'action du gouvernement je voudrais là encore évoquer plus précisément un service qui contribue de manière importante, bien que méconnu, à la sécurité des Français, je veux parler du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale l'ESG DSN qui comprend entre autres l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, le centre de transmission gouvernementale et le Groupement interministériel de contrôle, la montée en puissance de ces services est réel, nous la saluons néanmoins ils demeurent en deçà de leurs homologues britanniques ou allemands, tant en terme d'effectifs que de moyens, la problématique du recrutement notamment est crucial, comme l'illustre la compétition que doit livrer Lancy avec des géants du web pour attirer les talents dans le domaine de la cybersécurité nous estimons que notre effort de défense passe également par le renforcement de ses agences qui nous permettent de mieux combattre les nouveaux types de menaces en 1er ne lieu la menace cyber. Sous réserve de ces quelques interrogations portant surtout sur les crédits dédiés aux juridictions administratives et au service de détente de défense rattaché au 1er ministre le groupe les indépendants républiques et territoires votera les crédits de ses missions.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, un mot sur le budget de l'Élysée qui a quand même animé les débats à la fois à l'Assemblée et est 3 millions, 3 millions sur 100. Est ce qu'il s'agit de construire une piscine olympique, dans les jardins de l'Élysée, est ce qu'il s'agit de construire un terrain de badminton dans les Terres anglaises, non, on sait de quoi il s'agit, il s'agit de renforcer la sécurité du président et de son entourage, vous connaissez le contexte, il s'agit de la mise en place de la cellule de coordination des services de renseignements et il s'agit en fait d'améliorer la protection des systèmes informatiques et nous savons tous comment ces choses-là se passent, on a vu ça aux États-Unis, La députée de France insoumis The qui a dénoncé le fait, je cite, que le président de la République puisse se servir dans la caisse, ce son expression, je pense que c'est un propos qui est outrage et à la limite de la diffamation, je sais qu'un nouveau cas budgétaire est en préparation, où doit être mise en place, peut-être Monsieur le Ministre, vous pouvez nous en dire un mot, je passe sur le la, la Cour de justice de la République sur le conseil et contrôle de l'État, moi je me réjouis du renforcement des moyens de la Cour nationale du droit d'asile, c'est quelque chose derrière lequel nous courons depuis des années, 54 emplois vont permettre à cette juridiction d'augmenter le nombre de de cas traités et de réduire, alors j'ai probablement pas les mêmes chiffres que Monsieur Kanner, on me dit de 13 à 6 mois le délai moyen d'instruction des évidemment Sophie évidemment le nombre de demandes entre-temps temps augmentent de façon extrêmement forte, c'est quelque chose sur lequel nous avons longtemps demandé des moyens nouveaux et, plus largement, je souscris à la proposition du rapporteur spécial de l'Assemblée nationale, monsieur Daniel, la baronne, qui est le député d'Indre-et-Loire et donc quelqu'un de tout à fait respectable qui consiste à évaluer l'impact des réformes apportées aux procédures contentieuses en matière de droit des étrangers, les juridictions financières restent restent stables, pas de commentaire à faire, et enfin, je voulais demander vous demander, monsieur le Ministre, quel était le degré d'avancement de la certification des comptes des collectivités locales qui étaient en cours sur le du Conseil économique, social et en environnementale, bon, on va voir ce qui se passe, puisque il y a une grande réforme qui est payé, il est prévu d'en faire une sorte de Holding think tanks comme on dit, peut-être de lui donner des moyens supplémentaires et peut-être faudra-t-il revoir la dotation je me réjouis de voir que les effectifs de l'Anssi augmente de 25 ETP chaque année entre 2018 et 2022, c'est quelque chose, nous savons tous, c'est très important, le degré de menace des cyber attaques est important et nous Français de l'étranger, nous en savons quelque chose puisque nous avons été privés du droit de vote électronique aux élections législatives parce que l'y dit s'est déclaré en situation telle qu'il ne pouvait pas garantir le le produit qu'ils étaient en train d'élaborer enfin je me réjouis de l'achèvement de l'opération de restructuration de l'îlot Fontenoy Sigurd et je constate avec satisfaction que son enveloppe budgétaire est resté à peu près dans les les lignes qui qui avait été fixé le regroupement d'une grande partie des services du 1er ministre et des autres, plusieurs autorités indépendantes au sein de ce centre de gouvernement va permette de dégager d'un d'indispensables économies de fonctionnement loyer ma salariale etc, d'après le bleu budgétaire les immeubles naguère occupé par les entités qui ont emménagé dans les bâtiments Séguret Fontenoy devraient être vendus en 2018, monsieur le Ministre, pouvez-vous nous indiquer à combien est évalué le montant prévisionnel de ces cessions immobilières, la subvention la hausse de la subvention accordée à la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT qui porte le nom de deal dire pas pas le le mieux qu'on est trouvé, c'est comme ça, ces moyens supplémentaires lui permettront notamment d'assurer pleinement ses nouvelles missions en matière de lutte contre l'et LGBT phobies et contre le les actes d'antisémitisme dont on voit que malheureusement il perdure dans notre pays, voilà donc pour toutes ces raisons, notre groupe, le groupe de la République en marche votera ces crédits.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre Madame messieurs les rapporteurs mais, chers collègues, l'examen des crédits budgétaires de ces 3 missions traduit une très grande stabilité par rapport à la loi de finances pour 2017. S'agissant de la mission, pouvoirs publics, ces crédits n'augmente que de 0,0 8 pourcent entre 2017 et 2018, c'est donc une quasi-stabilité le budget des 2 assemblées parlementaires et donc stabilisé, comme c'est le cas depuis maintenant 5 ans 518 millions pour l'Assemblée nationale et 324 millions pour le Sénat, soit près de 84 pourcent des crédits de la mission seul progresse finalement à hauteur de 3 pourcent la dotation de la présidence de la République. Au-delà de ces chiffres, l'enjeu est ici celui de l'efficacité de la dépense publique et du bon fonctionnement de notre Parlement ni démagogie, laquelle affaiblirait nécessairement à la représentation nationale ni gabegie, c'est la seule voie sur laquelle. S'engager pour rétablir la confiance et le lien de nos concitoyens avec la représentation nationale. S'agissant des crédits budgétaires de la mission, les contrôle de l'État, il progresse de 2,2 pourcent cette année un rythme analogue à celui de l'an dernier où les crédits avaient été relevés de 2 pourcent. L'augmentation est porté pour les 3 quarts par le programme 165 retraçant les crédits de juridiction administrative et en particulier par la Cour nationale du droit d'asile pour amortir la hausse de plus de 30 pourcent du contentieux de l'asile 51 emplois sont ainsi créés auprès de la CNDA. La question du maintien au sein de la mission du programme 340 relatif au Haut Conseil des finances publiques reste posée, se pose surtout Monsieur le Ministre, la question de l'indépendance des chevaux au Conseil des finances publiques vis-à-vis de l'administration. Dans son audit de juin dernier, la Cour des comptes a en effet montré que l'évaluation des hypothèses du recettes et de dépenses par le Haut conseil rester tributaire des informations communiquées par les services de Bercy. La création d'un organisme indépendant sur le modèle britannique favoriserait la sincérité de textes budgétaires présentées au Parlement, favorisant du même coup la qualité de nos débats. Est elle envisageait, Monsieur le Ministre, s'agissant enfin de l'ami. C'est en direction de l'action du gouvernement les moyens budgétaires son temps alors stabiliser 1,48 milliard d'euros de crédits de paiement en hausse très légère de 0 26 Les priorités sont d'abord financés par des mesures d'économie, ce dont nous nous réjouissons. L'effort engagé lors des presque des exercices précédents dans les domaines de la sécurité du renseignement et de la cyberdéfense et prolongée, les effectifs sont ainsi rehaussés. De 18 équivalents temps plein selon nous nous réjouissons. Que l'effort budgétaire soit ciblée sur la sécurité et les services de renseignement est une très bonne chose sur le triennal 2018, 2020 la mission contribuer à la performance et à la main. C'est de la dépense publique or compte d'affectation spéciale pension ces crédits diminuent de 1 pourcent en volume. Vraiment, là, nous nous en félicitons, cette efficacité se traduit tout particulier tout particulièrement par la mise en place du projet immobilier Fontenoy figure qui permettra de mutualiser les fonctions support de l'ensemble des services du 1er ministre le détail de ce projet est désormais documenté début 2018 la plateforme accueillera 22 entités dont 2 secrétariats d'État, le gain escompté de ces mutualisation est estimé à 7 millions d'euros à ses efforts d'économie contribue également les autres, les autorités administratives indépendantes, malgré l'augmentation globale de leur crédit de 2 millions d'euros, cette nuance n'a toutefois pas vocation à être renouvelé, puisqu'elle doit seulement permettre aux autorités administratives indépendantes d'assurer l'organisation d'états généraux citoyen. De la révision prévue en 2018 des lois de bioéthique de 2011, compte tenu de leur cohérence globale, le groupe Union centriste votera les crédits de ces différentes missions, je vous remercie de votre attention.

Une entrée fracassante, monsieur le président, monsieur le Ministre Mesdames et messieurs les rapporteurs, chers collègues, j'ai l'honneur de porter la parole du groupe socialiste, sur les 3 missions d'importance que nous examinions ce matin, elles sont d'importance, parce qu'elle touche souvent à l'État dans ce qu'il a de plus noble de plus noble, mais pas forcément toujours de plus populaire auprès des citoyens, l'Élysée, les assemblées, les cours des comptes, les autorités administratifs, le Conseil économique, social et environnemental autant d'institutions indispensable à la République, qui mériterait parfois réforme, je le concède, mais des institutions dans lesquelles les agents publics ne renâcle pas la tâche, je tacherai donc d'être juste et bienveillant pour leur rendre hommage, je commencerai par la mission, conseil et contrôle de l'État, le groupe socialiste votera les crédits prévus Kanner a su nous convaincre de la pertinence de l'augmentation des crédits dévolus aux programmes, Conseil d'État et autres jus de réduction administrative et Cour des Comptes et autres juridictions financières, le renforcement des effectifs de la Cour nationale du droit d'asile qui fait face à une hausse importante du nombre des entrées enregistrées et la nécessité de pourvoir les emplois prévus pour les juridictions financières constituent des objectifs que nous partageons tous, en ce qui concerne la mission, pouvoirs publics, je salue ici Jean-Pierre Sueur je ne me hasarderais pas à polémiquer sur les moyens prévus pour la sécurité du président de la République, cela a été dit avant moi ou ceux prévus pour l'activité de sa compagne, ces dépenses sont justifiées à l'Élysée, toujours, on ne peut que se féliciter de la volonté affichée de vouloir contenir le poste le déplacement, notamment en ce qui concerne les déplacements à l'étranger j'invite cependant l'exécutif à ne pas renier sur les crédits de climatisation, je salue la volonté de mettre en concurrence plusieurs prestataires pour l'engagement des dépenses prévues pour les voyages officiels, nous imaginons que le président de la République ne souhaite pas être accusé de privilégier telle ou telle agence de communication toujours dans la mission, pouvoirs publics, je note la baisse de 1,1 pourcent de la dotation pour Public Sénat, elle démontre un souci de bonne gestion, a salué dans la période de débats actuel sur l'utilité de la préservation de 2 chaînes parlementaires distinctes le budget du Conseil constitutionnel sera en baisse en 2018, en l'absence d'élections à contrôler, je relève d'ailleurs, même si je n'ignore pas la complexité de la tâche et l'augmentation du nombre de recours cette année que certaines décisions sur des recours d'importance se font toujours attendre en cette fin d'année 2017. En ce qui concerne la mission Direction de l'action du gouvernement j'ai dévoré le rapport de monsieur Leconte concernant la réforme de l'État, un des aspects de la mission Direction de l'action du gouvernement monsieur Leconte Revel avec beaucoup de précision que l'inflation législative n'est pas forcément la conséquence d'une logorrhée verbale sénatoriales on ajoutera à ses remarques sur l'importance prise par les articles additionnels issues d'amendements gouvernementaux, l'existence d'amendements gouvernementaux en catimini par des parlementaires, le problème n'est peut-être pas dans la lenteur du travail parlementaire et législatif, contrairement à ce que beaucoup veulent nous faire croire, c'est même peut-être l'inverse : je n'ai pas la sensation que les parlements du monde travaille mieux que le nôtre et la volonté d'aller vite, contribue, sous tous les gouvernements, quelle que soit l'étiquette politique à légiférer mal il faut alors trouver des cordes de rappel, ce qui est normal quand on est 1er de cordée avec un amendement gouvernemental voir avec un amendement gouvernemental porté par l'homme, un parlementaire s'il s'avère que le rapporteur du projet de loi fait les gros yeux au cabinet du ministre-au rythme de travail plus serein nous permettrait sans doute d'éviter ce genre d'père mais non, il faut aller vite et pourtant même les députés en marche, constate qu'ils n'ont plus le temps de réfléchir, autre exemple de la manière dont l'enfer peut-être pavée de bonnes intentions, monsieur Leconte à relever les difficultés dans l'application du décret du 18 mai 2017 sur la limitation du nombre de conseillers par cabinet des conseillers parlementaires mais pas les vôtres, pas ici, monsieur le ministre m'ont indiqué avoir des difficultés à me répondre en invoquant la petite taille des cabinets, alors je ne leur jette pas la Pierre, même si leur excusez difficilement audible, mais j'ai participé à des débats où je voyais bien que le ministre n'avait pas de réponse précise préparé, j'imagine que les taux du décret de mai 2017 finira par se desserrer, il paraît même selon un hebdomadaire satirique qui les contourner et si c'est le cas, je m'en félicite, je veux revenir pour terminer sur le cas de quelques autorités indépendante le CSA un budget stable mais pourrait voir ses prérogatives augmenter si l'on en croit le discours du président de la République de samedi dernier, je ne suis pas certain de partager le point de vue du président de la République sur une telle évolution du rôle du CSA mais je ne demande qu'à être convaincu, j'ai pu constater la dernière lors d'une mission effectuée pour le compte du précédent gouvernement que si certains membres ou salariés du Conseil disposait du bagage nécessaire pour aborder les questions numériques, ils avaient aussi à batailler en interne pour gagner en légitimité quel serait le fondement juridique d'une telle évolution de son rôle, le CSA contrôle des contenus télévisés en échange de la mise à disposition des fréquences, mais quelle serait la logique concernant Internet, je ne peux pas croire que le président Macron soutient une nationalisation de l'espace de liberté que constitue Internet peut-être souhaite-t-il suivre l'exemple chinois concernant enfin le défenseur des droits, j'ai bien pris connaissance des éléments sur les fonctions support mais je dois vous avouer que je m'étonne de la baisse que connaît l'Autorité dirigé par Monsieur Toubon, je n'ai pas été particulièrement actif ni défendu sa nomination mais je dois bien reconnaître qu'il incarne à merveille ce rôle de défenseur des droits le CSA voit son budget maintenu mais le défenseur des droits doit lui faire des efforts supplémentaires pourraient vous Monsieur le Ministre, éclairer la représentation nationale sur ce point, vous l'aurez compris le groupe socialiste votera les crédits pour les 3 missions que nous étudions. Bien, merci, la parole est maintenant à monsieur Christophe Castaner, secrétaire d'État auprès du 1er ministre chargé des relations avec le Parlement, vous avez la parole monsieur le ministre. Merci monsieur le président, messieurs les rapporteurs spéciaux madame qui a fait fonction de rapporteur spécial pour l'occasion, monsieur rapporterait Madame, rapporteur pour avis, mesdames, messieurs les sénateurs, 10 minutes pour tenter de répondre à l'ensemble de votre question est un exercice difficile et j'ai bien entendu l'invitation de Jean-Pierre Sueur a retrouvé des usagers, notamment ceux de Robert Badinter, mais permettez au modeste secrétaire d'État que je suis, de ne pas oser cette comparaison, surtout quand on sait que Robert Badinter a fini son engagement politique sur vos bancs au Sénat et donc l'ancien député que je suis ne nos aurait même pas osé cette référence là je vais tenter de répondre aux questions posées, mais seulement à celles sur lesquelles je peux apporter des éléments de réponse et je commencerai partira Madame Assassi, par exemple, que je ne me prononcerai pas sur, je cite la faiblesse des moyens dévolus aux chambres au Sénat et à l'Assemblée, tout simplement parce que nous sommes sur des sujets où votre indépendance implique effectivement que le gouvernement par compétences liées ne se prononce pas sur ces sujets-là, je voudrais vous remercier de la qualité de vos travaux de la modération de vos propos parce qu'effectivement, nous sommes sur des sujets aussi sérieux que le bon fonctionnement de l'État et donc il nous faut sur ces questions, pouvoir balayer la réalité de ce que nous vivons, et notamment pour les dotations aux pouvoirs publics, les crédits se caractérise, vous l'avez dit, par une grande stabilité par rapport à l'exercice précédent, est toutefois je rebondis tout de suite sur la question de l'augmentation des moyens dédiés à la présidence de la République, chacun l'a rappelé quand vous avez exprimé ce sujet Monsieur Richard Yung en particulier Jean-Pierre Sueur aussi en évoquant l'effort financier sous la présidence de François Hollande qui mérite effectivement d'être souligné, chacun a rappelé les 3 millions de crédits supplémentaires sont dédiés à la sécurité physique du président et de ses proches, de ses collaborateurs, mais aussi de la sécurité numérique parce qu'elle est essentielle et je crois que cela va dans le bon sens mais il est essentiel que nous puissions sur ces sujets comme sur d'autres faire toute la transparence et monsieur le sénateur Richard Yung m'a interpellé sur sa transparence accrue qui se décline à la fois par la charte de la transparence relative au conjoint du chef de l'État mais aussi avec l'adoption, conformément au rapport de la et aux préconisations de la Cour des comptes, d'un nouveau cadre budgétaire et comptable qui va transposer à la présidence de la République, les règles de la gestion budgétaire et comptable public de droit commun tout en tenons compte de la spécificité du pouvoir public constitutionnel s'agissant du Conseil constitutionnel sa dotation est quasi stable par rapport à 2017 et d'importantes préciser ça parce que certains se sont interrogées sur une baisse, mais la baisse n'était que mais pas et Jean-Pierre Sueur a rappelé pourquoi cette dotation hors dépenses exceptionnelles liées aux augmentations 2016 et 2017 pour préparer les campagnes présidentielles et les contrôles sur ces campagnes présidentielles et législatives font qu'aujourd'hui on est sur une légère augmentation, toutefois, ça a été dit, l'augmentation du nombre de questions prioritaires de constitutionnalité doit effectivement être entendu parce que ça implique aussi des moyens, une ingénierie une expertise supplémentaire s'agissant de la Cour de justice de la République une dotation est inscrite au PLF afin de lui permettre d'instruire et de juger les requêtes qui lui sont adressées, mais chacun sait effectivement qu'une évolution constitutionnelle est envisagée, nous verrons sa réalité, il y a une question concrète sur les coûts fixes de la CJR notamment les locaux dans lequel elle est installée il y a une réflexion en ce moment qui est conduite pour imaginer qu'elle puisse rejoindre les locaux du tribunal de grande instance dans l'île de la cité, c'est à l'étude, je réponds à tout dépendra en fait au fond de la réforme constitutionnelle à laquelle vous participerait bien évidemment j'en viens maintenant à la mission, conseil et contrôle de l'État, s'agissant des juridictions administratives l'objectif et beaucoup d'entre vous le rappeler, reste la maîtrise des délais de jugement les crédits augmentent d'un peu plus de 2 pourcent car quand une l'augmentation extrêmement forte des recours devant, là encore, vous l'avez dit la Cour nationale du droit d'asile, il nous faut et ça a été rappelé par Didier Rambaud par Patrick Kanner faire face et la création de 51 emplois lui sont destinées à cette évolution, et nous pensons effectivement que ce sera tendu et difficile mais en même temps 51 51 51 créations d'emplois, c'est non négligeables, je pense aussi qu'il faut avoir en tête, certains d'entre vous l'a rappelé que la dématérialisation des procédures, a permis grâce par exemple à l'application de télé recours d'économiser 4,5 millions d'euros de frais de justice depuis 2013 le recours obligatoire à la médiation préalable doit aussi et les nouveaux outils procéduraux qui existé et que nous allons développer Davos aussi permettent de faire des économies substantielles sur ce sujet, en ce qui concerne les juridictions financières, les dépenses ont maîtrisé les dépenses de personnel augmentent très légèrement, je n'ai pas balayer tout ce qui a été dit évoquer encore par Patrick Kanner et Richard Yung, je pense que il est important qu'on puisse s'appuyer sur ces juridictions, notamment pour l'expérimentation de la certification des comptes des collectivités territoriales, cela est évoqué, il faut monter en puissance sur ce sujet-là, 25 collectivités expérimentatrice ont été sélectionnés l'expérimentation se déroulera jusqu'en 2023 faut en l'évaluer et en tirer tous les enseignements nécessaires sur la question du positionnement du Haut Conseil des finances publiques et certains d'entre vous ont évoqué Madame Julien Monsieur Rambo, je voudrais vous dire que le gouvernement est favorable à l'idée que le Haut Conseil des finances publiques soient rattachés dans le cadre des procédures qui existent sur les juridictions financières, je ne doute pas de la capacité de cette autorité d'avoir tous les moyens de contrôle sur l'état et je ne doute pas de sa capacité à les utiliser et à dire ce qu'il pense sans difficulté et aujourd'hui personne ne peut douter de leur indépendance, sur ce sujet, un mot encore sur le Conseil économique, social et environnemental vous dire parce que la question a été posée, que les travaux sont, comme pour le Sénat, l'Assemblée nationale, placée sous l'autorité de leur président respectif en lien avec la ministre garde des Sceaux, des réflexions sont en cours, celles sur le CESE ont bien avancé en interne au 16 le président Bernasconi, m'a demandé un rendez-vous ce matin pour mener présenter et nous aurons certainement l'occasion d'en parler tous ensemble, j'aborderai pour terminer la mission Direction de l'action du gouvernement à titre liminaire, je précise qu'un amendement présidente présenté par le gouvernement et adopté à l'Assemblée, a procédé à une minoration de 3 millions d'euros des visas à eux et des crédits de paiement or titre 2 pour prendre en compte et là il y a eu des augmentations, les conséquences des décisions annoncées lors du rendez-vous salarial du 16 octobre les crédits de cette mission sont stables en valeur par rapport à la loi de finances 2017, un certain nombre de mesures nouvelles sont prises en compte et beaucoup d'entre vous ont parlé de la mutualisation dans l'opération immobilière se goure Fontenoy constitue un bel exemple il y a des économies substantielles affaire est faite dans ce cadre-là, elles sont évalués de lors de 3,5 millions d'euros par an, mais elles sont importantes aussi en terme d'effectifs, certains d'entre vous, moi, interrogé sur la situation du défenseur des droits, dont on pouvait penser qu'il perd 3 équivalents temps plein à la lecture statistique des chiffres ou comptable, la réalité c'est qu'il dégage 4 équivalents temps plein supplémentaires pour me Z pour mener à bien les missions nouvelles qui lui sont confiés, c'est lié justement à cette économie de moyens de fonctionnement fait sur l'ensemble du site qui lui permet de dégager cela. à terme, nous pensons que nous pouvons globalement économiser 52 équivalents temps plein que 7 sites seront libérés à la suite de l'emménagement à Ségur Fontenoy qui pourraient être vendus et la question m'a été posée par le sénateur Delfau, le sénateur Young pour un montant évalué à environ 160 millions d'euros de recettes pour l'État, parmi les mesures nouvelles inscrite au PLF figurent un renforcement de la sécurité, beaucoup d'entre vous, moi, interpellé sur ce sujet et sénateur qui a dit que le compte sont sur ces sujets très mobilisés, vous avez raison, c'est un sujet majeur, je voudrais évoquer là encore les crédits consacrés à la coordination de la sécurité et de la défense qui progresse de 3 pourcent en 2018 avec de nouvelles créations d'emplois, 15 au GIC ça été rappelé par le sénateur moisir 25 à Lancy, certains trouvent ces chiffres insuffisant, j'ai entendu Olivier quasi que espéré plus mais c'est non négligeables quand même sur ces questions, il est important de noter quand même que l'agence a vu ses effectifs passer de 122 équivalents temps plein, à 2009 à 540 équivalents temps plein fin 2017, l'objectif du plafond dans le est à 685 équivalents temps plein en 2022, j'ai entendu les inquiétudes qu'on peut être exprimée sur les conséquences de ces créations d'emplois sur les fonctions depuis support du

dans les métiers du numérique et des systèmes d'information, une circulaire du 1er ministre du 21 mars 2017 a posé les grands axes du plan d'action dans ce sens, soyez plus généralement rassurer et assuré que le gouvernement est pleinement conscient des efforts en matière de 6 coeurs IT de systèmes d'information, cela doit être poursuivie amplifiée, notamment par un renforcement de la gouvernance de la cyber quelle sécurité au sein des ministères ou le développement d'une politique d'achat, la mieux adaptée possible s'agissant des fonds spéciaux, il a été dit qu'ils étaient en baisse, ça n'est pas le cas, l'augmentation est très légère de quelques centaines de milliers d'euros mais il se situe aujourd'hui à 67,38 millions d'euros pour mémoire en 2015, ils étaient à 49,4 millions d'euros. Je vais balayer rapidement vu, j'ai déjà dépassé mon temps de parole, ce que je voulais évoquer avec vous, c'est peut-être un mot si vous m'y autorisez monsieur le président, sur la 1000 cas madame de scène a évoqué effectivement et d'autres sénateurs ont évoqué cela, c'est un sujet évidemment important, je suis comme vous attacher à la forfaitisation je dis ça, c'est plus facile que contraventions analyse à Sion il y a toujours le risque de se tromper sur ce mot, c'était un engagement du président de la République, le Sénat l'avait porté en 2011 en 2015 les rappeler : nous souhaitons que cela puisse venir en discussion vite et notamment de prendre en compte cette aborder la situation particulière de nos départements d'outre-mer qui sont particulièrement frappés par ces conduites addictives, mais il y a l'alcool ou liés à la drogue sur lequel il faut un énorme travail de prévention, ça a été dit, évidemment je vous rejoins sur ce sujet, je vais, si vous le permettez, je ne pourrais pas répondre à tout, sinon je vais être trop bavard évoquer aussi la conscience et l'importance que nous accordons aux moyens pour les autorités administratives indépendantes, je pense à la Cada ou au CIC, elles ne je pense aussi à la CNIL, qui a été évoqué par Tina Turner Jean-Yves Leconte qui doit faire face à un nouveau cadre européen avec une double évolution à la fois un règlement une directive sur lequel nous faudra être mobilisés, je pense aussi au CSA, vous l'avez évoqué le président de la République souhaite lui donner ou élargir ses missions, il faudra travailler sur cet objectif et je compte sur les travaux sénatoriaux pour nous y aider et nous accompagner, je terminerai mon intervention a été crédits du problème 333 qui sont consacrés à l'immobilier au fonctionnement de nos services territoriaux l'qui progresse de 1,4 cette progression est notamment due à une harmonisation progressive des prestations d'action sociale dans les services déconcentrés harmonisation financé à hauteur de 5 millions d'euros pour nos agents pour nos personnels qui font face au quotidien émission toujours délicate qui mérite d'être accompagné, je voulais saluer, mesdames, messieurs, pour clore mon propos, je crois que vous avez dit les uns et les autres, la réalité de ce que sont ces Budgets qui nous sont présentés, ils sont difficiles parce que les missions sont difficiles mais ils correspondent à cet objectif de maîtrise de la dépense publique est essentiel et qui doit tous nous mobiliser, mais en même temps qu'doivent permettent de décliner des priorités parce qu'effectivement, il s'agit pas de reconduire à l'identique ou de rajouter un ou ou 2 pourcent chaque année au budget pour penser qu'on gère bien notre pays, mais plutôt d'assumer un certain nombres de choix pour faire face aux exigences de nos concitoyens, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie. Merci, merci, Monsieur le Ministre, donc nous allons maintenant procéder au vote des crédits de la mission, pouvoirs publics, figurant à l'État B il n'y a pas de d'explications de vote puisque tout le monde a utilisé son son temps de parole en introduction préalables. Donc je mets jamais au voile les crédits de cette mission, qui est pour.

je mets au les crédits de cette mission, qui est pour. Qui est contre. Toujours 3, merci donc les crédits sont adoptés. Vote des crédits de la mission Direction de l'action du gouvernement qui est pour. Qui est contre. Je pose question personne proteste qui s'abstient. donc une abstention. Donc, maintenant, on vote, donc ils sont adoptés, nous allons procéder au vote, donc des crédits du budget annexe publications officielles et information administrative, il y Donc, qui est pour. Qui est contre. Et il s'abstient. L'abstention donc ces crédits sont adoptés, je vais suspende la séance, elle sera reprise à 14 heures 30 pour l'examen de la mission santé puis de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances se réserve d'avoir achevé l'examen de ces 2 missions, nous pourrions ensuite examiné la mission défense à partir de 18 heures 30, la séance est suspendue.